j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Raymond Tarcy, qui fut sénateur de Guyane de 1980 à 1989.

Monsieur le président, monsieur le vice-président de la commission, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour aborder les enjeux relatifs à la vie associative,

Le texte qui nous réunit cet après-midi traite d'un sujet majeur pour les structures associatives : leur trésorerie. Comme le consacre l'adage, « l'argent est le nerf de la guerre » ; cela est d'autant plus vrai s'agissant d'associations dont les ressources sont, pour la grande majorité d'entre elles, limitées et complexes à obtenir et à élargir. Cette conviction, nous l'avons tous ici ; je la partage, en tant que secrétaire d'État chargé de la vie associative, mais aussi en tant qu'élu local, puisque, à mesure que les forums des associations se succèdent chaque année, nous prenons le pouls de ce qu'est aujourd'hui la réalité de la vie associative dans notre pays. Nous avons lancé plusieurs chantiers pour développer et diversifier le financement des associations ou pour les aider à accroître leurs ressources. Je pense aux annonces que j'ai faites dans le cadre de ma feuille de route, que j'ai présentée le 29 novembre dernier, sur les groupements d'employeurs pour faire des économies d'échelle, ou sur le plancher de dons à 10 000 euros, pour favoriser le mécénat des TPE et des PME dans les territoires, au plus près des organisations, dans une logique de synergie territoriale. Cette proposition de loi intervient directement dans le cadre de ces chantiers et de cet objectif. Elle a notamment pour objectif de lever les freins à la constitution de fonds propres par les associations, leur permettant d'investir ou de se projeter dans le plus long terme- nous savons combien c'est important également pour objectif de leur permettre de recevoir leurs subventions dans des délais qui correspondent aux réalités de gestion quotidienne d'une association, et d'une structure en général. Elle a pour objectif, enfin, de leur permettre de profiter, par le biais du fonds pour le développement de la vie associative, le FDVA, notamment, des fonds bancaires associatifs inactifs, et donc non utilisés aujourd'hui ; ce sujet revient régulièrement dans le débat depuis maintenant plusieurs années. fait suite à un travail de longue haleine mené par l'ensemble des acteurs associatifs. Le Mouvement associatif a travaillé pendant un an à un rapport qui a été remis au Premier ministre il y a maintenant plus d'un an. Ce rapport, ensuite repris par un certain nombre de groupes politiques, m'a moi-même aidé à nourrir la feuille de route que j'ai présentée le 29 novembre dernier. Les mesures qui se retrouvent dans ce texte font directement écho à ce rapport du Mouvement associatif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce texte a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Ce vote était important ; c'est un vote en faveur des associations et du développement de leur action dans les territoires, jour après jour, de répondre aux attentes et aux besoins sociaux : animer le périscolaire, gérer un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mener des actions culturelles pour tous les âges,

Les associations sont indispensables à la vitalité de notre pays ; leur assurer des facilités complémentaires pour développer et gérer leur trésorerie, c'est participer à cette indispensable action. Les deux ans qui viennent de s'écouler ont entretenu des doutes, des inquiétudes, parfois des critiques, dans le monde associatif, que la fin des emplois aidés a cristallisés. Cette mesure était essentielle, car il n'est pérenne pour aucune structure de bénéficier d'une forme de subventionnement déguisé, au travers d'un emploi, alors que les ressources ne sont ni stables, ni récurrentes, ni variées. Il faut penser la solidité et la pérennité des modèles associatifs en favorisant la diversification des ressources, des modèles d'organisation, des modèles économiques et des modèles de gouvernance, ainsi que le travail collaboratif, toutes ces mesures permettant une véritable structuration et un développement robuste.

continuer à le faire en poursuivant la simplification des demandes de subvention et la hausse progressive des conventions pluriannuelles d'objectifs qui sécurisent les ressources des associations. très forte qui vient des associations : elles veulent plus de prévisibilité pour ce qui concerne leurs ressources. Nous y travaillons, nous avons commencé à y travailler s'agissant de la politique de la ville, et nous poursuivons ces travaux qui nécessitent évidemment une coordination avec les collectivités locales. L'article 1 de cette proposition de loi a été supprimé en commission. Je le regrette ; c'est pourquoi je demanderai, au nom du Gouvernement, son rétablissement. Il permet en effet aux associations de conserver les excédents raisonnables liés à une subvention publique. Cette disposition permettrait très concrètement de renforcer des logiques de performance sans rien renier de la mission d'intérêt général portée portée par les associations. Cela leur permettrait également de renforcer leurs fonds propres, leur donnant les moyens, demain, d'investir et de développer leurs actions sur les territoires, dans une logique, toujours, de prévisibilité et de prospective. L'article 1 , quant à lui, visait à instaurer un délai maximal pour assurer le versement des subventions publiques. La discussion autour de ce délai a été l'occasion d'échanger avec un certain nombre d'associations d'élus d'élus des territoires, qui partageaient l'idée qu'il est nécessaire de donner de la visibilité aux associations et de se fixer des objectifs réalistes. Ce délai de soixante jours, donc, a été discuté avec les associations d'élus ; son instauration donne de la visibilité et sécurise l'action des associations au plus près des citoyens tout en préservant un délai de paiement réaliste et raisonnable, à la fois pour l'État et pour les collectivités locales. L'article 2, qui n'a pas été modifié en commission, porte une mesure indispensable pour la simplification de la vie des associations, en leur permettant de réaliser des prêts à taux zéro entre structures d'un même groupement d'employeurs ou d'une même fédération. Il s'agit aussi d'une mesure d'incitation à la mutualisation des compétences et des ressources. Cette mutualisation est un levier majeur pour le développement du monde associatif

de la concrétisation du premier emploi, dont on sait qu'il est souvent une marche très difficile à atteindre pour des structures associatives. L'article 3 concerne l'analyse rendant possible la récupération des fonds des comptes bancaires associatifs inactifs, au bout de trente ans, passent dans le budget général de l'État. C'est là un serpent de mer, qui revient régulièrement, s'agissant du financement de la vie associative. L'an passé, ce sont 1,9 milliard d'euros de comptes bancaires inactifs qui ont été versés au budget général. Quelle part de ce montant relevait de comptes d'associations qui avaient été laissées en déshérence ? Nul ne le sait, puisque le tri et l'analyse ne sont pas faits aujourd'hui. Il y a dans ce montant une part

est l'enjeu, très important, de cet article 3. L'article 3 est né d'une très forte attente des parlementaires. Nous en avions parlé longuement, ici, dans le cadre de l'examen d'autres textes et de la procédure budgétaire : il s'agit en effet de prévoir la présence des parlementaires dans les commissions départementales du fonds pour le développement de de la vie associative. Ces commissions paritaires regroupent les représentants de l'État, des collectivités et des associations ; désormais, elles pourront intégrer des parlementaires. Il s'agit en définitive de se caler sur le même format que celui des commissions relatives à la dotation d'équipement par parallélisme des formes, mais aussi et surtout dans l'objectif d'assurer une représentation garantissant le maintien du caractère mixte de ces commissions. La diversité des regards et des expertises est indispensable pour faire les choix les plus pertinents possible pour les territoires. L'article 4 consistait, quant à lui, à permettre aux seules structures associatives reconnues d'intérêt général et fondations reconnues d'utilité publique de bénéficier de la mise à disposition d'un bien immobilier dont la propriété a été transférée à l'État, ce que l'on appelle communément les biens mal acquis. La commission du Sénat y a ajouté des organismes qui ne sont ni sous statut associatif ni reconnus d'intérêt général. J'entends les arguments qui ont été développés ; nous pourrons en discuter tout à l'heure. Mais j'ai la conviction que cet ajout éloigne de l'objectif d'aider prioritairement les associations. Je vous proposerai donc d'adopter un amendement visant à revenir à l'écriture initiale de cet article, pour rester dans un périmètre d'action De la même manière, je vous proposerai de réintégrer l'article 4 , supprimé alors qu'il ouvrait à toutes les structures associatives et fondations la possibilité de ne pas faire l'objet d'un droit de préemption, ce qui leur assurerait une sécurité juridique forte, s'agissant notamment des dons immobiliers qu'elles pourraient recevoir. L'article 5, que vous n'avez pas modifié- je vous en remercie -, porte sur l'évaluation de la fiscalité liée aux dons ainsi que sur le modèle économique des organismes d'intérêt général, qui repose majoritairement sur la générosité.

bénéficier de ces mesures, qui améliorent leur trésorerie. C'est aussi, selon moi, un enjeu pour les parlementaires de pouvoir être présents dans les commissions départementales du fonds pour le développement de la vie associative

d'autres perspectives. Je pense à la proposition de loi en faveur de l'engagement associatif, dont nous avons déjà débattu ici ; je pense au projet de loi de finances et à d'autres vecteurs qui pourront nous rassembler. Je souhaite donc que nous puissions avancer, toujours dans l'optique de faciliter la vie quotidienne de nos associations, qui en ont besoin, et surtout de renforcer le lien social et la vie démocratique de notre pays, qui a besoin de ces associations partout sur le territoire. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations, dont nous discutons aujourd'hui, a été adoptée par l'Assemblée nationale le 26 mars dernier. Elle est issue d'une proposition de loi de Mme Sarah El Haïry, qui a ensuite été nommée rapporteure de la commission des lois de l'Assemblée nationale, et de plusieurs membres du groupe MoDem. Composée initialement de six articles, elle a été considérablement réécrite et étoffée en séance publique à l'Assemblée nationale elle se composait de dix articles avant son examen par la commission des lois du Sénat. Nous sommes tous attachés au monde associatif et nous avons conscience du rôle de plus en plus important qu'il joue dans la vie de nos communes. Simplifier la gestion des associations et alléger la tâche de ceux qui s'y consacrent est évidemment un objectif partagé. Aujourd'hui, c'est la commune qui est le premier partenaire des quelque 1,5 million d'associations actives que compte notre pays, et il existe un réel lien de confiance entre collectivités et associations. La commission des lois a cherché à préserver ce lien en refusant de faire peser sur les collectivités territoriales des contraintes excessives qui risqueraient de le fragiliser. Il est vrai que la relation entre collectivités et associations a évolué au cours des dix dernières années. Les subventions aux associations ont baissé, tout comme les dotations aux collectivités. Pour autant, collectivités et associations continuent de travailler ensemble, généralement en bonne intelligence. La commission a supprimé l'article 1, qui inscrivait dans la loi l'obligation de prévoir, dans les conventions signées entre l'autorité administrative et les associations qui perçoivent une subvention, les conditions dans lesquelles l'organisme à but non lucratif peut conserver un « excédent raisonnable » sur les ressources non utilisées. Cette notion d'excédent raisonnable, à vrai dire très mal définie, vient du droit européen. à l'origine à une simple faculté. Elle s'inscrit dans le cadre très particulier du régime des subventions, qui ne sont pas considérées comme des aides d'État par les instances de l'Union. En pratique, les collectivités peuvent donc déjà, en droit, laisser une part des subventions non consommées aux associations. Ce que prévoyait l'article 1 de la proposition de loi allait au-delà, en reconnaissant implicitement un droit à la conservation de subventions publiques sans tenir compte de la réalité des collectivités territoriales. La commission a considéré que cette disposition imposait une contrainte supplémentaire aux collectivités dans leurs relations avec les associations, sans pour autant garantir que ces dernières auront de l'argent à conserver.

À l'instar des délais de paiement applicables aux contrats de la commande publique, le délai de paiement pour l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements est fixé à soixante jours à compter de la notification de la décision d'attribution ou,

Aucune collectivité ne peut verser en une seule fois une subvention de plusieurs dizaines, voire centaines, de milliers d'euros, comme semble le prévoir le texte de l'article 1 . Les collectivités doivent avoir la possibilité de gérer dans le temps les subventions qu'elles versent, car elles-mêmes reçoivent leurs dotations de manière fragmentée, et de plus en plus tardivement. Inscrire dans la loi une obligation que les collectivités ne pourront pas toujours honorer paraît mettre inutilement en cause leur responsabilité et celle de l'État. La commission a adopté sans modification les articles 2 et 3 de la proposition de loi, même si, à titre personnel, je m'interroge sur leur portée et sur leur intérêt. Après débat, la commission a maintenu l'article 3 , qui tend à permettre la participation des parlementaires aux collèges départementaux de la commission régionale du fonds pour le développement de la vie associative. Cette mesure est justifiée par le fait que ce FDVA bénéficie d'une dotation qui relevait auparavant de la réserve parlementaire il s'agit de donner aux députés et sénateurs un droit de suivi sur ces sommes. C'est là, à mon sens, un bien maigre palliatif à la suppression de la réserve parlementaire, dont pouvaient bénéficier certaines associations. En effet, les montants alloués aujourd'hui sont largement inférieurs à ceux dont les associations bénéficiaient dans le cadre de la réserve parlementaire, ce qui les pénalise. La commission a été favorable à l'article 4, qui entend inscrire dans la loi la possibilité de confier à des associations d'intérêt général ou à des associations et fondations reconnues d'utilité publique la gestion d'immeubles saisis lors de procédures pénales.

au profit des organisations non lucratives, et donc à instaurer une restriction du droit de préemption des communes. Cette disposition a un passé législatif tortueux, et je tiens à saluer le travail

La commission a estimé que, si une collectivité décide d'user de son droit de préemption, par ailleurs très encadré, sur un bien qu'elle entend utiliser pour un projet, il n'est pas illégitime qu'elle puisse acquérir ce bien, même dans le cas d'un legs à une association, fondation ou congrégation. Elle a donc supprimé cet article. L'article 5 consiste en une demande au Gouvernement d'un rapport sur la fiscalité des dons et legs et sur les moyens de développer et de promouvoir la philanthropie. L'Assemblée nationale travaille déjà sur cette question, et ce rapport interviendra dans ce cadre. La commission a adopté les articles 5, 5 et 5 de la proposition de loi, et l'ensemble du texte ainsi modifié. Incontestablement, plusieurs des mesures de ce texte peuvent être utiles aux associations. D'autres D'autres ne sont pas acceptables, selon nous, car, malgré l'importance des associations dans la vie de notre pays, elles ne sauraient être placées par la loi au même niveau que les collectivités territoriales.

Vive la République ! » : c'est par ces mots que les sénateurs conclurent leurs débats lors de l'adoption du projet de loi relatif au contrat d'association, le 22 juin 1901. Quoi de plus républicain, en effet, qu'une loi qui, consacrant la chose publique, combinait l'objectif de laïcisation tel qu'il était recherché à l'époque et la liberté d'association, dans un contexte de peur des congrégations ? Quoi de plus républicain qu'une loi mettant fin à un interdit de 110 ans, celui de constituer des groupements professionnels et de se syndiquer ? Ce cadre, établi grâce à l'habileté de Pierre Waldeck-Rousseau, a résisté à l'épreuve du temps et reste aujourd'hui le socle de la vie associative française. Nos associations sont le creuset de notre vie sociale, le rempart face à l'individualisme croissant aussi, je souhaite rendre hommage aux 16 millions de bénévoles que compte ce pays, ces femmes et hommes qui ne comptent pas leurs heures et n'exigent rien en retour. Disons-le : l'objectif de cette proposition de loi déposée par le groupe MoDem à l'Assemblée nationale est louable, et notre commission, grâce au travail de sa rapporteur, a simplifié un texte qui, sur certains aspects, revenait à imposer des contraintes supplémentaires à nos collectivités.

conséquence, modifié les pratiques des collectivités, qui auraient dû faire face à la difficulté de définir avec chacune des associations la hauteur de cet excédent raisonnable. Reconnaissons qu'il y a plus simple.

Se posera sans doute le problème du non-recouvrement, mais, si un tel cas de figure devait se présenter, le droit commun ferait loi. Nous approuvons également les mesures visées aux articles 3 et 3 . La transformation par l'Assemblée nationale de la disposition censurée de la loi Égalité et citoyenneté permettant l'affectation du produit des comptes bancaires d'associations en déshérence gérés par la Caisse des dépôts et consignations au fonds pour le développement de la vie associative est une bonne chose. Toutes les associations ne roulent pas sur l'or ; chaque initiative susceptible d'améliorer leur quotidien et de leur permettre d'offrir davantage de services ou de mener plus d'actions doit ainsi être encouragée. Plus surprenante, mais tout aussi appréciable, est l'ouverture aux parlementaires de la participation aux collèges départementaux de la commission régionale du FDVA. Ce droit de regard accordé aux parlementaires prouve peut-être que la réserve parlementaire avait toute son utilité et n'était pas, comme nous avons pu l'entendre à l'époque, « un mécanisme venant entretenir le soupçon du clientélisme ». Ça, c'est sûr ! Deux ans après sa disparition, aurait-on quelques doutes sur une décision teintée de démagogie ? À vrai dire, ce qui nous interroge, dans ce texte, c'est qu'il tend à s'appliquer à toutes les associations, sans distinction. L'équilibre proposé par Waldeck-Rousseau, dont je faisais l'éloge au début de mon propos, est peu à peu dévoyé la distinction entre les associations de droit commun et les associations cultuelles instaurées par loi de 1905 s'est peu à peu effacée. Dans certains cas particuliers, comme celui d'associations cultuelles ayant pris la forme de la loi de 1901, la question du financement public est problématique, ce financement étant en totale contradiction avec la loi de 1905. loi de 1905. Oui ! Cette situation devient absolument inacceptable lorsque les exonérations fiscales permises par l'article 200 du code général des impôts dépassent le montant des subventions accordées. Il s'agit d'une entorse frontale à l'interdiction de financement des cultes. Un peu de cohérence législative serait nécessaire sur ces sujets. Bravo ! En adoptant l'article 4 tel quel, nous permettrions à l'État de mettre des locaux saisis à la disposition d'associations ou fondations cultuelles, certes reconnues d'utilité publique, mais assurant malgré l'exercice et l'enseignement d'un culte. Aussi proposons-nous- tel est le sens de l'amendement que nous avons déposé à cet article -de supprimer l'article 4 de la loi de 1907, qui permet aux associations de type loi de 1901 d'assurer l'exercice d'un culte à titre dérogatoire. Il est prévu que les associations concernées aient jusqu'à juillet pour changer leurs statuts et devenir ce qu'elles auraient toujours dû être : des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905. J'entends bien que ce que nous vous proposons ici demanderait un débat plus large. Mais c'est un signal que de nombreux membres de mon groupe, attachés au principe de séparation des Églises et de l'État, souhaitaient envoyer, dans la perspective des futurs débats sur la laïcité-

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je vais emboîter le pas de la collègue qui m'a précédée en vous parlant moi aussi des associations cultuelles. Puisque les associations sont des associations, qu'il s'agisse de pêche à la ligne ou de gestion des lieux de culte, il se trouve que la loi est la même pour tout le monde. Si, donc, favoriser le financement des associations est un objectif extrêmement louable, il ne faut pas être naïf pour autant, et je voudrais, à ce titre, faire quelques observations. Le financement des associations ne peut aller sans transparence. Je sais bien que le travail parlementaire est un travail de répétition ; je vais donc répéter ce que j'ai déjà dit plusieurs fois à cette tribune. Le dernier rapport de Tracfin contient cette année encore un chapitre entier intitulé « Renforcer la transparence des associations à but non lucratif », relevant des carences dans le fonctionnement du secteur, tout autant que le manque de transparence dans la gestion de certaines associations.

Il en est ainsi des obligations comptables au premier euro de financement public. Il en va ainsi de la création d'un fichier comportant éventuellement le nom des trésoriers et présidents d'association.

ma chère collègue. Bref, il y a des marges de progrès, et j'espère que le Sénat adoptera les amendements que je défendrai tout à l'heure.

les associations sont des acteurs majeurs de la vie publique. Elles contribuent à l'activité sociale, économique, culturelle, patrimoniale et écologique de nos territoires. Constitué de plus de 1,5 million d'entités, le monde associatif est indispensable dans l'animation de nos villes et de nos campagnes. Il compte environ 2 millions de salariés, soit 5 % du salariat national, pour un volume financier de 110 milliards d'euros. Les associations sportives, mais aussi les associations d'insertion ou d'aide, comme le réseau Aide à domicile en milieu rural, créent des liens sociaux solidaires dans nos territoires. Ce ne sont pas moins de 16 millions de bénévoles qui agissent, sans être rémunérés, donc, pour l'intérêt général et le bien d'autrui.

Toutes ces personnes consacrent donc gratuitement de leur temps. Elles doivent être soutenues. Il faut apporter plus de souplesse à leur fonctionnement. Tel est l'intérêt que nous voyons dans cette proposition de loi. Je souhaite tout particulièrement saluer à cette tribune le travail de ces bénévoles, leur engagement et leur dévouement, qui est admirable. Il est naturel que les pouvoirs publics soient des partenaires pour nos associations. Le versement de subventions est la juste reconnaissance de leur contribution dans la mise en oeuvre des politiques publiques sur nos territoires. Ces dernières années, la réduction de la dotation globale de fonctionnement a mis en péril le monde associatif, associatif, victime par ricochet de la diminution des moyens financiers dont disposaient les collectivités locales. La trésorerie des associations est ainsi devenue un enjeu important, leurs fonds propres étant généralement trop faibles, ce qui constitue un frein à leur capacité à innover dans la mise en oeuvre d'actions ou de projets. En ce sens, l'article 1 de la proposition de loi déposée par notre collègue députée Sarah El Haïry constituait une avancée nécessaire. Il devait permettre aux associations de conserver légalement un éventuel excédent trop versé au-delà d'un bénéfice raisonnable, dans la définition de la subvention. Je le rappelle, un excédent doit finalement être restitué. En effet, les associations disposent en général de peu de fonds propres, ce qui peut constituer un obstacle à leur fonctionnement. Cette situation est liée à leur modèle économique, non capitalistique, et à la nature de leurs activités, essentiellement à but non lucratif. Dans le cadre de la relation avec les financeurs publics, des solutions peuvent être trouvées pour faire reconnaître et appliquer le principe d'excédent raisonnable. Cet excédent consiste à conserver une partie des fonds octroyés dans le cadre d'un financement public, pour autant que les objectifs partagés aient été atteints et que l'excédent constitué relève d'une maîtrise des dépenses n'ayant pas nui à l'exécution des missions. Pour ces raisons, j'ai déposé un amendement visant à rétablir l'article 1. Dans la même optique, l'article 1 venait répondre aux besoins de trésorerie des associations. En effet, les associations, notamment les plus petites, peuvent, lorsque la subvention qui leur est attribuée est versée tardivement, faire face à des difficultés de trésorerie. Aussi, cet article avait pour objet d'encadrer les délais de versement des subventions. À l'instar des délais de paiement applicables aux contrats de la commande publique, le délai de paiement pour l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements était fixé à soixante jours à compter de la notification de la décision d'attribution ou, le cas échéant, de la survenance de l'événement prévu par la convention portant attribution d'une subvention. J'ai donc déposé un amendement visant à rétablir l'article 1 , supprimé par la commission des lois du Sénat, mais en modifiant toutefois le délai de versement des subventions par rapport à la version issue de l'Assemblée nationale : quatre-vingt-dix jours au lieu de soixante jours, laissant ainsi plus de souplesse pour les collectivités. Il me semble que c'était l'un des points litigieux. Enfin, je regrette que l'article 4 ait été supprimé par le Sénat en commission des lois sous prétexte qu'il contrevenait au droit de regard des communes et instituait une restriction du droit de préemption des collectivités, sachant qu'elles ont toujours le droit de faire une expropriation. Les donations constituent une source importante d'apports pour les associations et les fondations. À titre d'exemple, entre 2013 et 2015, 35 % des fondations reconnues d'utilité publique ont une dotation allant de 500 000 euros à 17 millions d'euros. Dans de nombreux cas, les immeubles apportés à la dotation sont ceux qui permettent la réalisation de l'objet social de la structure. L'ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations avait exclu les biens de ces dernières du champ du droit de la préemption urbaine. Or la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a récrit un article du code de l'urbanisme avec pour effet involontaire de faire disparaître cette mesure et de soumettre de nouveau ces biens au droit de préemption. Un amendement avait été présenté et adopté en première lecture du projet de loi Égalité et citoyenneté au Sénat. Toutefois, pour des raisons de forme, le Conseil constitutionnel l'avait censuré. L'article 4 , introduit à l'Assemblée nationale, visait donc simplement à corriger les effets de cette suppression malencontreuse. C'est pourquoi j'ai déposé un amendement tendant à le rétablir. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les chiffres concernant le secteur associatif sont éloquents. Les associations sont très présentes dans les territoires. Elles contribuent au maillage de notre cohésion sociale. L'État et l'administration n'ont pas vocation à tout faire. Il est heureux que des femmes et des hommes agissent avec l'élan du coeur pour mener à bien des actions qui témoignent que, vivre en société, c'est aussi se prendre en charge sans systématiquement se tourner vers la puissance publique. Les représentants associatifs sont des personnes motivées, qui constituent un vivier d'interlocuteurs indispensables pour les élus locaux, nous aidant ainsi à répondre au mieux aux attentes des habitants de nos communes. À notre tour, montrons-leur de la solidarité face aux Il faut conclure, mon cher collègue. Les associations peuvent également constituer des leviers économiques et font vivre le tissu économique local. Elles animent la vie de nos territoires et des quartiers de nos villes. Veuillez conclure ! Les associations ont besoin de souplesse, et non de contraintes

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en France, le Mouvement associatif fait preuve d'une vitalité exceptionnelle. On estime à 1,3 million le nombre d'associations en activité, au sein desquelles sont engagés 16 millions de bénévoles et 1,8 million de salariés. Chaque année, 70 000 associations nouvelles se créent. Dans mon département, où l'on compte plus de 2 000 associations, l'engagement citoyen est également très actif. Le « travail »- je mets des guillemets à dessein -qu'accomplissent les associations est remarquable, qu'elles oeuvrent dans les secteurs culturel, sportif, sanitaire ou social. Elles créent du lien social, assurent le relais de l'État et des collectivités, et pallient malheureusement parfois leurs défaillances. Je parle en connaissance de cause, car mon engagement en politique a été fortement motivé par mon expérience dans le milieu associatif. En 2003, face à la problématique encore naissante de l'exclusion des plus jeunes à Mayotte et à l'absence de prise en charge par les institutions,

Le 28 janvier 2015, j'inaugurais le seul et unique établissement de placement éducatif de l'île, appelé, c'est-à-dire la « maison de l'espoir » si vous avez bien suivi la leçon de shimaoré, afin de répondre à la problématique des mineurs sous main de justice répondant au dispositif de l'ordonnance de 1945. Voilà pourquoi je considère, à titre personnel, que la présente proposition de loi de nos collègues députés du groupe MoDem, qui nous réunit aujourd'hui, est particulièrement importante pour les associations. Elle s'intéresse à un sujet fondamental pour leur fonctionnement : leur trésorerie. Les quatre mesures qu'elle contenait initialement, issues du rapport du Mouvement associatif remis au Premier ministre le 9 novembre 2017, elles-mêmes issues du rapport du Haut Conseil à la vie associative de 2014, répondaient à des revendications anciennes et légitimes du monde associatif. L'Assemblée nationale était parvenue au vote de ce texte à l'unanimité. Je dis bien « à l'unanimité » ; c'est suffisamment rare pour être souligné. C'est la raison pour laquelle je regrette que, lors de son examen en commission des lois, le Sénat soit revenu sur certaines de ces avancées et compromette au sein de notre Haute Assemblée un tel consensus. Je pense notamment aux suppressions de la possibilité pour les associations de conserver l'excédent raisonnable d'une subvention et de la mise en place du délai de soixante jours pour le versement des subventions, qui nous apparaissent comme un véritable recul. L'argument selon lequel ces dispositions pourraient venir troubler les relations d'équilibre entre associations et collectivités ne semble pas pertinent, car celles-ci ne ne comportent aucune contrepartie coercitive pour les collectivités. Au demeurant, les associations d'élus n'ont pas manifesté le moindre désaccord depuis le mois de mars.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le million et demi d'associations que compte notre pays joue, grâce à ses 16 millions de bénévoles, un rôle essentiel dans notre société par les missions que ces associations assurent, depuis les actions de solidarité à destination des plus démunis aux activités sportives ou culturelles, en passant par des missions de service public dévolues à l'État ou même à certaines collectivités ; ensuite, par les valeurs qu'elles portent, celles du bénévolat, de l'engagement et de la solidarité, qui sont au coeur de notre pacte républicain ; enfin- plusieurs l'ont souligné -, par la place qu'elles occupent dans la vie économique de notre pays, avec presque 2 millions de salariés et un budget total de 113 milliards d'euros, soit l'équivalent de plus de 3 % du PIB. Soutenir ces structures, qui sont au coeur de la cohésion sociale et qui ne suscitent pas toujours l'intérêt et la reconnaissance qu'elles méritent, est donc indispensable. Cette proposition de loi vise à leur apporter un tel soutien en améliorant leur trésorerie, ce qui- vous l'avez noté à juste titre, madame la rapporteur -revient à tenter d'accroître leurs ressources. C'est indispensable tant les associations sont mises à rude épreuve ces dernières années. La diminution extrêmement importante des contrats aidés a été un coup d'une violence telle

pour des associations n'ayant pas forcément des reins assez solides. Effectivement, ces emplois comportaient, par définition, une forme de précarité ; à ce titre, ils n'ont jamais constitué la panacée pour nous. Mais on ne peut pas nier

sous silence. La fin de la réserve parlementaire, également évoquée par un certain nombre de collègues, n'a pas été compensée par un abondement du fonds pour le développement de la vie associative du même montant ni à destination des mêmes types d'associations. Cela a évidemment des répercussions sur les associations, en particulier les plus petites et les plus locales. La liste des mesures qui handicapent la vie associative est malheureusement longue.

la baisse du budget destiné à ces dernières. Enfin, et la chose n'est malheureusement ni nouvelle ni négligeable, la diminution des dotations des collectivités locales continue d'avoir d'importantes conséquences sur les subventions attribuées aux associations. Dans ce contexte, la commission des lois a fait le choix, regrettable de notre point de vue, de supprimer un certain nombre de dispositions favorables aux associations au motif qu'elles contraindraient les collectivités locales. locales. Certains articles étaient peut-être imparfaits. Ils mériteraient au moins d'être discutés, voire améliorés en séance publique. C'est en ce sens que, comme d'autres groupes, nous avons déposé des amendements de réintroduction des articles, certes un peu modifiés, en écho aux revendications que le monde associatif, dans sa diversité, porte porte depuis bien longtemps maintenant. La question du trop-perçu et celle des délais de versement des subventions sont essentielles pour les structures associatives sans pour autant, à notre sens, placer les collectivités territoriales devant des difficultés insurmontables, pour peu que l'on travaille à des solutions adaptées. Nous regrettons que, au lieu de considérer que les collectivités, comme les associations, font face aux mêmes politiques austéritaires et que les difficultés des unes se répercutent inévitablement sur les autres, on contribue, en quelque sorte, à les opposer, dans une logique de gestion de la pénurie. Certes, la pénurie est toute relative, puisque les choix de diminuer la dépense publique sont évidemment politiques. L'ambition première de cette proposition de loi est modeste, mais pertinente. Elle permet au fond de trouver des sources de financement et de faciliter le fonctionnement budgétaire des associations sans avoir besoin de dégager énormément de ressources supplémentaires. Malheureusement, la suppression des articles 1, 1 et 4 rend cette proposition de loi encore plus modeste. En revanche, l'article 3 permettra d'avancer vers une proposition portée, là encore, depuis longtemps par le monde associatif : récupérer les fonds dormants des comptes inactifs des associations. Je ne sais pas si c'est un « serpent de mer », monsieur le secrétaire d'État, mais voilà en tout cas une occasion à ne

dernier. Rien que pour cela, la présente proposition de loi mériterait d'être votée. Mais, vous l'aurez compris, notre groupe souhaite profiter du débat en séance publique pour continuer de défendre les propositions du monde associatif qui avaient donné lieu à ce texte et qui nous semblent conserver toute leur pertinence, tant elles constituent des avancées importantes dans la gestion quotidienne des associations. J'espère que nous nous retrouverons en ce sens, en faveur de nos associations. La parole

Malheureusement, des amendements déposés bien tardivement, madame la rapporteur, ont fait exploser l'esprit de consensus qui aurait dû nous animer sur un sujet comme le financement du secteur associatif.

affichée d'amplifier l'engagement dans notre pays ou, du moins, de simplifier la vie des bénévoles et de faciliter l'accès aux financements. Le fait que 16 millions de bénévoles fassent vivre cette démocratie au quotidien est une richesse exceptionnelle pour la France. Ces Français nous obligent, nous obligent, nous, responsables politiques, à être à leur hauteur pour que tout soit fait en faveur de ce don de soi. Je n'oublie pas les quelque 2 millions de salariés qui oeuvrent dans le secteur à but non lucratif. L'esprit de consensus que j'évoquais ne doit pas se traduire par un blanc-seing donné au Gouvernement. Cette proposition de loi doit être vue pour ce qu'elle est : un petit pas visant à prendre en compte les attentes d'un secteur associatif en difficulté. En reprenant des demandes du secteur, ainsi que des mesures validées sous le précédent précédent quinquennat, notamment certaines votées dans le cadre de cette fameuse loi Égalité et citoyenneté, mais censurées par le Conseil constitutionnel, la proposition de loi allait dans le bon sens avant son passage en commission. Il convient néanmoins de ne pas oublier que ce texte intervient dans un contexte de désengagement de l'État envers le milieu associatif.

Le secteur associatif, les réseaux de l'éducation populaire ou les clubs sportifs, en renfort du service public, de l'école notamment, doivent être soutenus pour irriguer l'ensemble des territoires et apporter par leur présence un cadre et des repères aux enfants et aux adolescents. C'est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 Et cela doit se traduire concrètement, en amenant les nouvelles générations à s'impliquer dans le secteur associatif. J'évoquerai la situation du service civique.

L'évolution du financement des associations se traduisant par le recul du financement public, la proposition de loi vise à leur accorder de nouveaux moyens permettant de diversifier leurs sources de financement. La part du financement public des associations représentait 51 % de leurs ressources en 2005. Cette part ne cesse de se réduire. En 2011, elle atteint 49 %. Les subventions publiques ont reflué de 34 % à 24 % des ressources.

Ce changement pourrait aller à l'encontre de la spécificité du modèle français d'engagement associatif, dont tous les acteurs de terrain ont conscience. Les associations créent un lien social précieux à la Nation, notamment dans les territoires ruraux et périurbains de la République, par le service complémentaire au service public. Cela a été évoqué. Le risque Le risque d'une baisse de l'activité du monde associatif en raison d'une diminution des financements est également celui de faire reposer sur l'État une partie des missions que ce secteur assume. On constate que les mesures fiscales des précédents budgets favorisent fortement l'épargne. Cela n'est pas critiquable en soi, mais on remarque que la traduction concrète de ces mesures est une baisse très importante des dons

La réforme a fait passer le nombre de foyers assujettis à cet impôt de 358 000 à 120 000, soit 66 % de foyers en moins, supprimant l'incitation qu'avaient de nombreux contribuables à faire preuve de générosité envers les fondations reconnues d'utilité publique. Cette baisse de la collecte auprès des particuliers fortunés doit être replacée dans le contexte d'une baisse générale de la collecte grand public en raison de la réévaluation du taux de contribution sociale généralisée, qui touche notamment les retraités. La CSG est un frein à la générosité collective.

nous faisons du surplace, voire, avec la suppression de l'article 1, nous avons reculé. L'article 1 est la traduction législative d'une proposition sur le financement privé du secteur associatif émise par le Haut Conseil à la vie associative depuis 2014

La droite sénatoriale, je le regrette, invoque des risques de tensions dans les relations que les collectivités territoriales entretiennent avec les associations, alors que c'est sur l'association intéressée que pèsera l'obligation de définir la notion d'excédent raisonnable en démontrant le niveau de fonds propres nécessaires pour assurer son bon fonctionnement.

Contrairement aux observations émises par Mme la rapporteur, les collectivités pourront toujours gérer dans le temps les subventions qu'elles versent dès lors que le délai de versement de soixante jours court à partir de la notification de la décision dont elles sont à l'origine. En aucun cas le dispositif n'impose le versement de la totalité de la dotation, ce qui risquerait de créer des distorsions de trésorerie des collectivités territoriales. Enfin, la suppression de l'article 4 nous interroge. Cet article avait pour objet de rendre inapplicable le droit de préemption aux immeubles cédés à titre gratuit à des fondations, des congrégations ou des associations ayant la capacité de recevoir ce type de libéralités. Les motivations apportées à l'appui de la suppression de cet article par la majorité de la commission des lois du Sénat sont inappropriées. Une fois encore, madame la rapporteur, vous entendez opposer le droit des collectivités territoriales et l'intérêt du monde associatif, alors que l'objet principal de ce dispositif vise à corriger les contradictions apportées par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances

Même si nous aurions préféré une grande loi pour le secteur associatif, nous n'oublions pas que ce dernier a grandement besoin de ces premières mesures. ! Je Je rappelle que l'Assemblée a adopté la proposition de loi à l'unanimité. Je lance donc un appel à mes collègues de la majorité sénatoriale pour qu'ils reviennent sur leur vote en commission, afin que nous puissions rétablir les articles tels qu'adoptés par l'Assemblée nationale et nous diriger vers un vote conforme.

quelque part la preuve. Nos concitoyens s'investissent avec ferveur dans la vie publique. Ainsi, un Français sur quatre est bénévole et un foyer sur deux fait des dons à une association. Nous pouvons en être fiers, comme nous le sommes de nos élus municipaux, dont, je le rappelle, 370 000 sont bénévoles. Ils sont les artisans de la citoyenneté. Ces forces vives permettent à tous de se rencontrer, à travers une passion commune, mais aussi des convictions. En effet, à l'évocation de ce statut, nous pensons spontanément aux associations caritatives, culturelles ou aux clubs sportifs. Mais leurs activités sont très variées. En tant qu'ancien maire, je peux affirmer que le tissu associatif est une véritable richesse pour une commune. Je souhaite profiter de cette tribune pour évoquer, devant vous, une association que nous connaissons peu : l'Association d'Aide Pénale. Elle a été créée en 1978 afin d'apporter son concours au traitement de la délinquance et de contribuer à l'insertion sociale. Avec le temps, ses missions se sont élargies, allant jusqu'à la médiation pénale en 1990, à la réparation pénale en 1993, à l'organisation de stages de sensibilisation à la violence en 2011 et, enfin, en 2012, aux stages de soutien à la parentalité. Au vu de ces missions, pouvons-nous véritablement parler d'association au sens commun du terme ? Cette association joue un rôle d'auxiliaire de justice puisqu'elle est agréée par des tribunaux et chargée de la mise en oeuvre de mesures ordonnées par des magistrats. Je souhaite ici démontrer que les associations pallient trop souvent les manquements de l'État. Ce dernier ne doit en aucun cas se défausser ni se satisfaire En ces temps où la menace terroriste pèse sur chaque événement, nous demandons de plus en plus aux associations d'assurer elles-mêmes la sécurité de leurs manifestations, notamment des entreprises spécialisées. Au-delà du coût, où est l'autorité de l'État ? Le général Bertrand Soubelet titrait un de ses livres : Rappelons que la liberté d'association ne vaut que si elle peut s'exercer. Ce texte entend encourager une « philanthropie à la française » et je m'en réjouis, car cela va vers plus de responsabilisation et une prise en main de la chose publique par nos concitoyens. Cependant, cette philanthropie ne doit pas faire oublier à l'État qu'il doit se reformer afin de réaliser de réelles économies. Comprenez que nous ne pouvons pas encourager nos concitoyens à financer davantage les associations et « en même temps »-pour reprendre une expression à la mode -ne pas réduire leurs prélèvements obligatoires lorsque ces associations prennent, prennent, d'une certaine manière, le relais d'une administration trop lourde. Nous évoquons souvent les doublons au sein des collectivités, mais nous pouvons et devons également nous interroger sur des doublons entre les institutions et les associations, car toutes, répétons-le, ont directement ou indirectement la même source de financement : nos concitoyens. Comme beaucoup ici, je souhaite un État délesté et fort là où il doit l'être. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le monde associatif a explosé. Il est désormais un acteur incontournable de la vie économique. Ses missions se sont multipliées. Là où aucune collectivité n'a la fameuse « compétence », ni parfois les moyens, pour répondre à certaines attentes et besoins de la population, le monde associatif, tel un petit soldat providentiel, se lève et propose ses services. Les associations, désormais, rendent des quasi-services publics : il est grand temps que le législateur leur facilite la tâche. Alors, quelle bonne nouvelle que ce texte, qui présente un caractère d'urgence ! Enfin, on se penche sur ce sujet. Si la complexité administrative devenait rédhibitoire, si le monde associatif renonçait, alors il n'y aurait plus personne pour relever le défi et faire vivre la pratique sportive, artistique, mais également l'humanitaire, le social, les associations environnementales, la défense des consommateurs, l'enseignement privé, les Ehpad associatifs, les fédérations, les oeuvres, les centres sociaux et autres services d'aide à domicile, qui sont parfois devenus les plus gros employeurs de nos territoires. Ce texte, entre autres dispositions, prévoit que les parlementaires puissent siéger dans les commissions d'attribution du FDVA. Nous connaissons la plupart de nos associations, nous connaissons leurs acteurs et leurs actions. En retrouvant une place légitime dans cette instance, nous participerons concrètement au soutien de ce maillage de nos territoires. L'article 3 propose également une mesure très intéressante. Nous connaissons tous, en effet, le cas des associations, qui, devenues « sans objet » ou ayant perdu leurs leaders, tombent dans un profond sommeil. Telle Blanche-Neige, elles attendent le baiser qui les ramènera à d'autres aventures. Elles gèlent des trésoreries qui seraient fort utiles à d'autres causes. Ces comptes dits inactifs pourraient être fléchés vers le FDVA. Il nous faudra seulement veiller à ce qu'ils ne s'égarent pas en route vers les gouffres sans fond d'autres déficits totalement étrangers à l'affaire. La mesure, par ailleurs, n'aura de sens que si elle vient s'ajouter aux fonds d'État fléchés chaque année vers le monde associatif, et non pas permettre un retrait discret des finances publiques devant l'arrivée de cette manne providentielle. Sans entrer dans le détail des autres dispositions, je dirai que, dans sa globalité, ce texte recevra le soutien du groupe Union Centriste, pour la souplesse et la dynamique qu'il apporte, pour son ouverture à la mutualisation et au secteur privé, la seule limite étant de ne pas apporter de contrainte supplémentaire aux collectivités. Pour aller encore plus loin, je souhaite profiter de l'occasion pour attirer votre attention, monsieur le secrétaire d'État, sur une proposition portée initialement par notre collègue Catherine Troendlé. Les associations sans but lucratif organisent un nombre toujours plus grand de manifestations, qui contribuent à l'attractivité de la vie locale. Pour ce faire, elles recourent bien souvent de façon ponctuelle à des aides de type gardiennage, manutention, service, entretien, etc. Pour tous ces emplois, et sans aucune dérogation, il faut réaliser, chaque fois, des déclarations à l'Urssaf, même pour un poste occupé quelques heures. Cette lourdeur administrative les étouffe. C'est pourquoi nous proposons, pour les associations à but non lucratif, une dérogation, dans la limite de six fois par an, à ces obligations déclaratives. Ce serait un simple alignement de la réglementation sociale sur la réglementation fiscale, puisque la loi exonère les recettes de six manifestations annuelles. Je vous remercie d'étudier cette disposition, qui entre parfaitement dans le cadre des débats de ce jour, raison pour laquelle je me suis autorisée cette digression. que nous croisons quotidiennement, de la plus petite jusqu'aux énormes vaisseaux, je réalise que tous les acteurs ont le même visage. Le visage de l'engagement, le visage de la passion pour une cause, le visage de mon voisin.

n'a les moyens humains et financiers de remplacer le monde associatif et son armée de bénévoles. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la France compte aujourd'hui 1,3 million d'associations et 13 millions de bénévoles. C'est une richesse extraordinaire. Je le mesure chaque jour dans mon département où il existe une réelle il existe une réelle dynamique associative. J'ajoute que le nombre de personnes souhaitant s'engager ne cesse d'augmenter. C'est une bonne nouvelle : cela veut dire que la France sait se montrer solidaire. Cette solidarité, il faut l'encourager, surtout dans une société où les rapports interpersonnels peuvent parfois être violents, où les repères de notre modèle démocratique sont bousculés, où le relativisme a cassé tous les repères existants et où l'individualisme est croissant. Tocqueville définit ainsi l'individualisme dans : il s'agit du « désintérêt pour les affaires publiques » et de « l'amour des jouissances matérielles ». Cet individualisme menace la responsabilité politique du citoyen à l'égard du bien commun. C'est ce contre quoi nous devons lutter et c'est ce que permet justement l'engagement associatif : bâtir une société plus solidaire, active, concrète, au plus près des réalités quotidiennes. J'imagine que nous partageons tous ce constat. Avec cette proposition de loi, qui vise à améliorer la trésorerie des associations, on ne peut s'empêcher de penser que le Gouvernement se lance dans une opération de séduction à l'égard du monde associatif.

Ainsi, en 2018, 47 % des associations déclaraient être inquiètes quant à l'évolution de leur situation financière. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, le Gouvernement a décidé de réduire drastiquement le nombre de contrats aidés. Entre 2017 et 2018, le nombre de ceux-ci, dans dans les associations, est passé de plus de 80 000 à une trentaine de milliers et 12 500 employeurs associatifs ont disparu en 2017.

Aujourd'hui, vous nous présentez un texte dont l'ambition principale est d'accompagner le développement des associations en leur permettant de renforcer leurs fonds propres et d'obtenir de nouvelles formes de financement. Cette initiative législative vise à pallier l'absence, à l'heure actuelle, d'un plan d'action du Gouvernement, pourtant initié il y a déjà plus d'un an. Elle reprend certaines préconisations du rapport du Mouvement associatif, remis au Premier ministre en mai 2019. Ainsi, toutes les mesures qui simplifient la gestion des associations et allègent la tâche de ceux qui s'y consacrent sont un objectif partagé. J'aimerais revenir sur ce qui a motivé les amendements de la commission des lois et la réflexion menée par notre collègue rapporteur, Mme Eustache-Brinio. ont été supprimés : il s'agit de ceux qui soumettaient les collectivités territoriales à des obligations de paiement ou à des limitations en matière de préemption manifestement excessives par rapport à la réalité des relations entre les associations et les collectivités sur le terrain. Ne faisons pas peser sur le dos des collectivités des contraintes supplémentaires. Je rappelle qu'elles sont déjà soumises à une insécurité financière, avec la disparition de la taxe d'habitation et, parfois, la poursuite de la baisse des dotations. Faisons, par ailleurs, attention à ne pas altérer la relation de confiance qui existe entre les collectivités territoriales et les associations.

votera ainsi le texte modifié par la commission et rappelle son soutien au monde associatif, si important dans la vie de nos territoires. Car c'est souvent dans le tissu associatif d'aujourd'hui que l'on trouve les citoyens engagés qui seront les élus de demain au service de la République. Très bien

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, un texte en faveur du monde associatif est toujours une bonne chose, surtout à l'heure où celui-ci est confronté à de graves difficultés financières. Je suis bien placé pour le savoir puisque j'ai codirigé, avec notre collègue Jacques-Bernard Magner, la mission d'information sur les conséquences de la baisse des contrats aidés De tout temps, la situation financière des associations a été une préoccupation, mais, depuis quelques mois, leurs difficultés de trésorerie se sont aggravées. C'est un vrai sujet d'inquiétude pour la pérennité de nos associations et de leurs actions. En effet, depuis le début de ce quinquennat, des signaux désastreux, d'une violence inouïe, ont été envoyés au monde associatif. La transformation de l'ISF, la hausse de la CSG, le prélèvement à la source ou bien encore les mouvements sociaux ont eu indéniablement, cela a été dit, une incidence sur la collecte de dons. La fin des contrats aidés- 459 000 en 2016 contre 100 000 attendus en 2019 -, la baisse des subventions publiques, la suppression de la réserve parlementaire et l'inadéquation du fonds pour le développement de la vie associative sont autant de coups fatals assénés au tissu associatif. Que dire de ce FDVA, mis en place par pur dogmatisme, qui devait être abondé à hauteur des sommes accordées à nos associations dans le cadre de l'ancienne réserve parlementaire, soit 120 millions d'euros, et qui ne l'est finalement qu'à hauteur de 25 millions d'euros ? Une fois de plus, le compte n'y est pas. Ce gouvernement fait des économies sur le dos du monde associatif alors que les besoins sont immenses. Continuer à faire mieux avec moins n'est plus acceptable. Je vous l'assure, monsieur le secrétaire d'État, les associations sont à l'os. J'en veux pour preuve la situation du FDVA dans mon département, le Vaucluse, en 2019. Il bénéficiait de 270 600 euros de crédits. Les services ont reçu des demandes de 191 associations à hauteur de 1 105 316

Les parlementaires que nous sommes, eux, le savent. Nous le mesurons au quotidien quand, dans nos départements, nous rencontrons ces bénévoles désespérés de n'avoir pu acheter de nouveaux maillots pour les équipes de jeunes ou de n'avoir pu transporter gratuitement les enfants au tournoi du village d'à côté. Nous mesurons aussi leur désarroi grandissant lorsqu'on leur demande d'être porteurs de projets innovants dans le cadre d'appels à projets de plus en plus complexes, tout en continuant de jouer un rôle pivot dans notre société. Je porte ce combat avec énergie, car je suis convaincu que l'altruisme de ces hommes et de ces femmes impliqués dans le quotidien des autres mériterait plus de reconnaissance et beaucoup plus de considération. C'est grâce à ces 16 millions de bénévoles que nos communes connaissent une vie culturelle, sportive et sociale particulièrement dense ; sans oublier, bien sûr, l'engagement de nos jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Ces hommes et ces femmes de bonne volonté sont souvent, aux côtés des maires, « les premiers de cordée », dans nos villages, dans nos quartiers. Personne ne peut se substituer au travail remarquable qu'ils effectuent au quotidien. Les remercier aujourd'hui est bien la moindre des choses et ce texte est aussi une façon de leur exprimer notre infinie reconnaissance. Cette proposition de loi, même si elle aurait pu être beaucoup plus ambitieuse, va dans le bon sens. En prévoyant diverses mesures financières de soutien aux associations, elle donne corps à plusieurs propositions que le Haut Conseil à la vie associative réclamait depuis plusieurs années. Il est primordial de renouer le lien de confiance avec les associations. J'espère que cette politique « du petit pas » y contribuera un peu. Car, il ne faut pas s'y tromper, elle ne corrigera pas totalement les signaux désastreux qui ont été envoyés au monde associatif depuis le début de ce quinquennat.

visibles ou crédibles aux yeux de leurs partenaires. L'article 1 visait à intégrer la possibilité pour les associations de conserver un éventuel excédent trop versé au-delà d'un bénéfice raisonnable, dans la définition de la subvention. En effet, bien que rien ne les empêche juridiquement de réaliser des bénéfices, les associations disposent en général de peu de fonds propres, ce qui peut constituer un obstacle à leur développement. Cette situation est liée à leur modèle économique, non capitalistique, et à la nature de leurs activités, essentiellement à but non lucratif. Dans le cadre de la relation avec les financeurs publics, des solutions peuvent être trouvées pour faire reconnaître et appliquer le principe d'excédent raisonnable. Il s'agit de conserver une partie des fonds octroyés dans le cadre d'un financement public pour autant que les objectifs partagés aient été atteints et que l'excédent constitué relève d'une maîtrise des dépenses n'ayant pas nui à l'exécution des missions. Tel est l'objet de cet amendement. En droit, ce qui n'est pas utilisé doit être restitué.

l'article 1 adopté à l'Assemblée nationale, qui vise à permettre aux associations de conserver et de reporter un bénéfice raisonnable sur une subvention qui n'a pas été entièrement

collègues, nous avons la possibilité d'adresser un signal fort aux associations en adoptant une mesure simple, qui leur permettrait de mieux fonctionner au quotidien, pour se développer, innover, investir et, finalement, remplir les missions d'intérêt général que nous-mêmes, en tant que décideurs locaux, nous leur confions bien souvent. L'ensemble des acteurs du secteur associatif partagent le même constat. Alors que nous étions sur le bon chemin après l'examen du texte par les députés et leur vote unanime,

possibilité : il permettrait aux seuls organismes à but non lucratif de conserver l'excédent d'une subvention non dépensé en introduisant la notion d'excédent raisonnable, afin de renforcer leur assise financière. Est-il sérieux de susciter de fausses peurs

pourraient entretenir avec le secteur associatif. Or, nous le savons, c'est dans une démarche de dialogue et de confiance que nous travaillons bien souvent et, heureusement, avec nos partenaires associatifs au niveau local. Ces partenaires doivent disposer de fonds propres afin d'avoir une visibilité budgétaire. Pour les acteurs locaux, cette bonne pratique existe déjà au quotidien sur le terrain. Nous savons que les collectivités continueront à exercer un contrôle vigilant, dans la confiance. Tel est l'esprit de cet amendement de rétablissement.

Comme cela vient d'être rappelé, cet article vise à intégrer la possibilité, pour les associations, de conserver un éventuel excédent de fonds octroyés dans le cadre d'un financement public, pour autant que les objectifs partagés aient été atteints et que l'excédent constitué relève d'une maîtrise des dépenses n'ayant pas nui à l'exécution des missions de l'association. Cet article est très important. Nous ne comprenons pas vraiment pourquoi Mme la rapporteur a voulu le supprimer, vidant ainsi le texte d'une grande partie de sa substance.

Les autoriser à conserver un excédent trop versé leur permettra de renforcer la trésorerie des associations, afin qu'elles aient les moyens d'investir et de développer leur action sur l'ensemble du territoire, dans le but de remplir leurs missions d'intérêt général. Dans sa version adoptée par nos collègues de l'Assemblée nationale, le champ d'application de cet article était limité aux seuls organismes à but non lucratif, c'est-à-dire à ceux qui souffrent le plus du manque de moyens. Cette proposition figurait déjà dans le rapport de 2014 du Haut Conseil à la vie associative sur le financement privé du secteur associatif. C'est une mesure que nombre d'acteurs du milieu associatif appellent de leurs voeux depuis plusieurs années. Ne leur donnons pas l'impression que la représentation nationale les oublie dans un texte qui les concerne au premier chef.

D'expérience, je sais qu'aucune collectivité ne met en péril l'avenir d'une association en lui reprenant les fonds dont elle a besoin. Donc, sauf à vouloir envoyer une espèce de signal politique aux associations, je ne vois pas l'intérêt de légiférer sur une pratique qui existe déjà de façon parfaitement naturelle et logique dans nos bassins de vie, entre les collectivités territoriales, que ce soient les communes, les départements ou les régions,

ce n'est pas le rôle premier du législateur. Son rôle premier est de faire la loi, d'établir des règles, si possible simples, claires, qui ne souffrent pas trop la contestation ou l'interprétation.

Toutefois, plutôt que de supprimer totalement la disposition, il nous semble qu'une légère adaptation du dispositif serait bienvenue. Ainsi, nous proposons que, à défaut d'un versement complet de la subvention, au moins le premier acompte soit provisionné dans les soixante jours suivant la notification.

Deuxièmement, l'engagement d'un versement complet ou partiel dans les soixante jours permet à la fois à la collectivité d'échelonner ses subventionnements, ce qui n'est pas rien, mais aussi aux associations de construire leurs projets au fil de l'eau. En effet, nous en sommes tous conscients, les associations doivent procéder à des achats au dernier moment. Quand elles se préparent en avance, elles trouvent d'autres sources de financement, qui entraînent des flux financiers et complexifient largement le contrôle du financement des associations. connaissons des associations dont les bénévoles avancent sur leurs fonds propres des achats et se font rembourser une fois la subvention versée. Dernière option, qui entraîne encore des flux financiers à rebours : les associations achètent à crédit. Troisièmement, il nous semble essentiel de le rappeler, les associations font une multitude de demandes de subvention pour chaque projet. Or, bien souvent, les différents échelons territoriaux conditionnent leur soutien à la participation financière d'autres collectivités, dans la limite des plafonds de financement public. De fait, lorsqu'une collectivité territoriale fait courir un très long délai entre sa notification de subvention et le versement de cette dernière, elle bloque parfois le processus pour d'autres collectivités et,,

que le délai soit raisonnable, il faut prévoir un délai de notification. Je dirais même que le délai de notification est peut-être plus important que le délai de versement, pour la sécurisation financière

Pour faire face aux délais trop longs de paiement, certaines d'entre elles ont recours aux cessions Dailly, mais cela suppose des frais bancaires qui fragilisent encore les trésoreries et qui peuvent poser des difficultés financières se répercutant sur l'ensemble de l'année. L'article 1 , inséré en séance publique à l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, répondait à ces difficultés, en inscrivant dans la loi un délai de paiement pour l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements. L'objectif de cet article était de faire en sorte que les subventions obtenues par les associations leur soient versées dans un délai raisonnable. Les communes garderont la maîtrise de leur budget dans l'attribution des subventions. Au regard de toutes ces considérations, il nous paraît pertinent d'encadrer les délais de versement des subventions, sur le modèle des délais de paiement applicables aux contrats de la commande publique. C'est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, de rétablir l'article 1 . Le délai, fixé à soixante jours à compter de la notification de la décision d'attribution ou, le cas échéant, de la survenance de l'événement prévu par la convention portant attribution d'une subvention, répond parfaitement à l'exigence d'un paiement rapide, et il convient à nombre d'associations.

bénéficient de dotations elles-mêmes très fragmentées et versées de plus en plus tardivement. Si l'on n'aide pas les collectivités à fractionner les subventions aux associations,

en termes de comptabilité publique. C'est une simple question de volonté et de bonne entente entre les dirigeants de l'exécutif de la collectivité locale et les associations demanderesses.

des bébés ne peuvent être vaccinés à temps, des personnes touchées par le cancer ne peuvent recevoir leurs médicaments, des malades de Parkinson peuvent être gravement atteints par la rupture de leur traitement. La liste est longue ... Face à ce constat, vous avez annoncé, madame la ministre, la volonté d'agir du Gouvernement. Pourtant, vos déclarations ne semblent pas montrer une volonté de s'attaquer à l'impuissance publique face aux laboratoires pharmaceutiques. Or ce point est majeur. Les laboratoires renchérissent les coûts en organisant les pénuries, prônent le recours aux flux tendus en réduisant les stocks pour maximiser les profits et délocalisent hors de France la production et la recherche.

Il est temps que tout cela change, que la filière pharmaceutique soit considérée comme stratégique et vitale, que l'État soit capable d'assurer l'approvisionnement de médicaments de qualité à des prix abordables. Que compte faire concrètement le Gouvernement pour atteindre ces objectifs ?

à mieux informer à la fois les patients et les professionnels afin de rétablir la confiance et la fluidité entre tous les acteurs. Le deuxième axe vise à mieux lutter contre les pénuries par de nouvelles actions de prévention et de gestion des risques sur l'ensemble de la chaîne de production et de distribution du médicament.

rassurer nos concitoyens : l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament, notamment les pharmaciens et les médecins, font aujourd'hui tout leur possible pour assurer la distribution des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Je les remercie sincèrement de leur implication. Le comité de pilotage permettra de rendre compte régulièrement de l'avancée de cette feuille de route. La parole

mais possessionnels -commis dans de nombreux cas par des hommes qui préfèrent leur femme morte plutôt que libre ; soixante-quinze femmes âgées de 20 à 90 ans tuées par la violence machiste. À la demande des associations et des familles de victimes, le Gouvernement, par votre voix, madame la secrétaire d'État, a annoncé un Grenelle des féminicides, qui se tiendra de septembre à novembre. La mise en commun des expériences sera bien évidemment utile. J'espère que, d'ici là, les conclusions de l'Inspection générale de la justice seront connues et que la même enquête sera menée dans les services de police et de gendarmerie. Toutefois, plusieurs décisions pourraient d'ores et déjà être prises, sans devoir patienter cinq longs mois supplémentaires. Ni la lutte contre les violences faites aux femmes ni la faiblesse des budgets pour les prévenir et pour protéger les victimes ne datent de mai 2017. J'en tiens pour preuve, madame la secrétaire d'État, que vous êtes chargée de mettre en oeuvre le cinquième plan triennal de mobilisation, ce qui veut dire que le premier remonte à quinze ans. ans. Le budget qui y est consacré, lequel avait pourtant augmenté de 50 % entre 2012 et 2017, n'a jamais été à la hauteur des besoins. Vous ne manquerez sans doute pas de me répondre que la hausse des moyens s'est poursuivie ces deux dernières années. Mais vous admettrez sans doute avec moi que les moyens ne sont toujours pas suffisants.

chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Je vous

de la question des moyens pour se pencher sur celle de l'effectivité des politiques publiques que nous mettons en oeuvre. Il faut véritablement que toutes les administrations, que les services de police, de justice et de gendarmerie sur les territoires puissent être engagés. C'est le sens de ce Grenelle. Tous les ministres concernés seront présents pour travailler et coconstruire avec les associations, les parties prenantes, les experts, les familles et les proches de victimes. Ce Grenelle sera conclu par le Premier ministre Édouard Philippe, pour arrêter ensemble un agenda concret et des mesures

La parole est à M. Claude Malhuret, pour le groupe Les Indépendants-République et Territoires. Nous désapprouvons la politique du ministre, vengeons-nous sur les élèves », voilà comment résumer la farce sinistre qui vient de se jouer dans nos lycées, transformés en ZAD- zones à délirer-par moins de 1 % de grévistes, condamnés par une condamnés par une grande majorité de Français et par une grande majorité de leurs collègues. Angéline, bachelière parmi beaucoup d'autres cités par, déclarait : « On a fait notre travail. Respectez-le et redonnez nos notes, ce n'est pas à nous de payer. Aujourd'hui, ce sont les élèves qui sont forcés enseigner la morale à certains de leurs professeurs. Le premier devoir des enseignants est celui de l'exemplarité devant leurs élèves. L'exemple que l'on veut donner aux enfants est-il celui de ne pas remettre ses copies ? Il ne viendrait jamais à l'idée des médecins d'arrêter de soigner les malades quand nous faisons grève ou même de ne pas remettre l'ordonnance. Les zadistes des salles d'examen en folie n'ont pas ces scrupules manque de respect envers les élèves, dont cette grève a tellement à coeur les intérêts qu'elle en fait ses premières victimes, manque de respect envers les familles qui leur confient leurs enfants, manque de respect envers leurs collègues, dont ils abîment l'image. Maintenant qu'ils ont perdu face à un ministre déterminé- ce qui n'était pas arrivé depuis des années-, ils dénoncent les inégalités. Mais qui a créé les inégalités entre les candidats si ce n'est les escamoteurs de copies ? Les mêmes annoncent déjà des préavis de grève en septembre. Ne pourraient-ils pas déposer un jour un préavis de travail ? On ne peut se permettre la réforme Blanquer », disent-ils. Mais peut-être l'éducation nationale ne peut-elle se permettre ces offusqués professionnels et leurs drôles de méthodes, qui auraient fait rougir de honte leurs ancêtres les hussards noirs. Monsieur le Premier ministre, je souhaite que vous nous assuriez de votre fermeté face aux révolutionnaires à statut protégé et de votre détermination à appliquer une réforme qui n'est pas seulement la réforme Blanquer, mais aussi celle de l'Assemblée nationale et du Sénat. La parole

Il a bien fait, et je lui apporte évidemment tout mon soutien, car nous devons faire en sorte que cet examen et ceux qui le passent soient respectés. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour dire

être opposée à tel ou tel aspect de la politique menée par le ministre de l'éducation nationale et le Gouvernement, mais qui considère qu'un enseignant doit transmettre un savoir et donner l'exemple.

Dans l'agglomération grenobloise, depuis plusieurs semaines, des actes communautaires viennent chaque jour fracturer un peu plus notre contrat républicain. À deux reprises, des femmes militantes, qui ont la volonté d'aller contre les interdits, ont fait le choix de défier l'autorité publique en venant se baigner en burkini dans les piscines municipales, qui est pourtant interdit par les règlements intérieurs. Dans le même temps, nous avons appris qu'une école salafiste que le ministre de l'éducation nationale a décrite comme « inspirée par des idéologies radicales » est toujours ouverte. Elle devait pourtant fermer, mais cette décision est suspendue dans l'attente d'un procès qui ne se déroulera pas avant novembre prochain. De telles situations illustrent une seule et même orientation qu'il faut dénoncer haut et fort : la fracturation communautaire de notre société, conjuguée à l'offensive d'une forme d'agression identitaire. Face à de tels actes, c'est notre pacte républicain qui chaque jour s'abîme un peu plus. Peut-on accepter que, tout l'été, la question du burkini se pose dans les piscines municipales ? Comment accepter qu'une école salafiste radicalisée puisse continuer d'accueillir des élèves lors de la prochaine rentrée ? Les élus locaux sont dans l'attente d'une réponse claire et stricte de l'État, afin de faire respecter sur l'ensemble du territoire la laïcité et les principes républicains de notre démocratie.

du principe de laïcité et de l'ordre public. Face à ce type de comportements, partout dans les quartiers victimes de replis identitaires et de communautarisme, qui en souffrent, nous avons lancé dans le cadre du plan interministériel de prévention de la radicalisation de nombreuses actions de contrôle de lieux,

L'ensemble de ces actes, nous le savons tous, n'a qu'un seul objectif : tester la République pour mieux la déstabiliser. Votre réponse doit être sans ambiguïté et de la plus grande fermeté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malgré les propos que vous venez de tenir. Nous sommes nombreux à appeler de nos voeux un débat sur la laïcité, afin de mieux la protéger et de la renforcer. Sans cela, vous laisserez perdurer, malheureusement avec une lâche complicité, un flou qui accentue les tensions dans notre pays.

Nous avons constaté que les chambres de métiers et de l'artisanat et certains directeurs de CFA réclament l'application de la réforme dès le mois de septembre 2019, soit à la prochaine rentrée scolaire. En effet, conformément au décret du 28 mars dernier, le paiement des CFA au « coût contrat » serait plus avantageux pour une majorité d'entre eux que l'ancien système dit des « coûts préfectoraux Madame la ministre, comptez-vous proposer aux CFA qui le souhaitent d'utiliser le nouveau système de financement dès la rentrée de 2019 ? Sinon, y aura-t-il une remise à plat en janvier 2020 pour tous les contrats antérieurement souscrits, afin qu'il n'y ait pas de distorsion financière entre anciens et nouveaux contrats ? L'État s'est aussi engagé à verser aux régions une enveloppe de 250 millions d'euros, au titre des dépenses de fonctionnement. Celles-ci pourront ainsi moduler territoire par territoire le taux de prise en charge des contrats et assurer le maintien de certaines formations en zone rurale. Rien n'est encore figé, a été faite d'un versement en octobre. Qu'en est-il exactement ? Les régions disposeront également de fonds d'investissement. Ces investissements doivent faire l'objet de conventions d'objectifs et de moyens conclues avec les OPCO. Le projet de loi prévoit que les critères d'attribution de ces fonds seront fixés par décret, après concertation

trois régions ont décidé de priver de trésorerie à la fin de l'année tous les CFA de leur région au moment de la transition. J'en appelle donc à l'intérêt général. On ne peut pas jouer avec les jeunes et les entreprises

iranien. Depuis quelques semaines, ce dossier suscite de vives préoccupations. Dimanche dernier, Téhéran a annoncé avoir commencé à enrichir son uranium

le rappelle, cet accord prévoit que l'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire en échange de la levée des sanctions politiques et économiques. Téhéran menace de prendre d'autres mesures si Paris, Londres et Berlin se comportent « de manière étrange ». D'une certaine façon, ces pays européens sont pris en otage par les positions extrêmes des États-Unis et de l'Iran. Cette crise est la conséquence directe du retrait unilatéral des États-Unis de l'accord de Vienne, effectif depuis 2018, et du rétablissement des sanctions économiques américaines, sans doute dans l'espoir de faire tomber le régime de Téhéran. L'économie iranienne est désormais en récession. en récession. L'initiative prise par l'Iran risque de faire voler en éclat un instrument essentiel pour la sécurité de l'Europe, de la région et du monde, même si la provocation américaine en est à l'origine. Face à cette crise, la France a déployé d'importants efforts diplomatiques, ce dont nous nous réjouissons. Hier, le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue américain. Il a également décidé dépêcher un conseiller diplomatique à Téhéran. Celui-ci est chargé d'« assembler les éléments d'une désescalade, avec des gestes qui doivent être faits immédiatement avant le 15 juillet », soit dans moins d'une semaine. Nous saluons cette initiative. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer

les faits que vous avez évoqués ont été constatés aujourd'hui par l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Iran a rompu deux reprises les accords de Vienne, à la fois par l'augmentation du stockage d'uranium faiblement enrichi, limité à 300 kilos, ainsi

Il y a des silences qui en disent long, comme il y a des paroles qui ne signifient rien. » Depuis le dépôt, en 2014, du dossier d'extension du plateau continental, le Gouvernement français est extrêmement silencieux sur ce sujet. Les propos tenus par Emmanuel Macron lors du grand débat à l'Élysée, en février 2019, ne nous ont pas rassurés. J'aimerais qu'on nous explique quelle est la stratégie de la France dans le cadre de la négociation de l'extension du plateau continental au large de Saint-Pierre-et-Miquelon.

vous m'interrogez sur la résolution du différend entre la France et le Canada s'agissant de la délimitation du plateau continental de la France au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous nos deux pays sont parties à la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Tous deux ont déposé un dossier de demande d'extension du plateau continental.

des litiges, la seule solution, pour la France, est de parvenir à un compromis bilatéral avec le Canada. À cette fin, la France a proposé en 2016 le lancement d'un dialogue d'experts franco-canadiens pour en discuter. Pour le moment, le Canada n'a pas souhaité entamer cette discussion, mais nous restons ouverts sur ce point. Sans attendre qu'une solution puisse être trouvée à ce différend, le Président de la République a évoqué récemment la question de Saint-Pierre-et-Miquelon avec le Premier ministre du Canada, lors des cérémonies du 6 juin, en vue de renforcer l'intégration régionale de l'archipel. Cette intégration renforcée doit pouvoir se matérialiser en particulier dans le domaine clé que le domaine de la pêche pour l'archipel. Au-delà du différend juridique entre la France et le Canada, la priorité du Gouvernement reste d'assurer le développement économique et social de l'archipel. Sachez, monsieur le sénateur, que Mme la ministre des outre-mer est particulièrement attentive à ce sujet. Nous avons l'occasion d'en parler très souvent pour essayer d'avancer. Mais, pour avancer, il faut être deux

Le Canada persiste à nier l'évidence et à refuser tout dialogue avec la France concernant le plateau continental, alors même qu'« il n'a pas hésité à trouver des solutions intelligentes avec d'autres États et partenaires en la matière », comme le rappelait Annick Girardin, députée à l'époque

Républicains. Au début du quinquennat, le programme Action publique 2022 était présenté comme l'alpha et l'oméga de la transformation de l'État. Il devait sortir le pays de l'ornière. Aux premiers jours de l'été 2018, nous vivions un psychodrame autour de la publication du rapport du comité Action publique 2022. Quatre mois plus tard, en octobre 2018, à l'occasion du second comité interministériel de la transformation publique, on apprenait que « près de 75 % des recommandations du comité se retrouvent dans les chantiers lancés par le Gouvernement Une telle rapidité et un tel taux de mise en oeuvre pour un rapport réputé écrit par des experts indépendants laissent pantois. En avril 2019, dans son programme national de réforme, le Gouvernement se félicitait des résultats obtenus Les transformations issues d'Action publique 2022 vont notamment se traduire par des baisses du nombre d'emplois publics, déjà mises en oeuvre par les lois de finances pour 2018 et 2019. » On aurait aimé y croire ! Malheureusement, ni la Cour des comptes ni la Commission européenne ne partagent votre autosatisfaction. En effet, la Cour des comptes, dans son rapport sur le budget de l'État en 2018, indique : « Bien que les créations de postes aient été très limitées par rapport aux trois années précédentes [ ...], la baisse nette des effectifs [ ...] prévue par la LPFP n'est pas encore engagée. Quant à la Commission européenne, sa lecture du programme de stabilité et du PNR 2019 est sévère. Permettez-moi de citer son avis du 5 juin : « Il n'apparaît pas clairement comment, et dans quels délais, ce programme de réforme contribuera par des mesures concrètes [ ...] à l'objectif très spécifique de réduction du ratio des dépenses au PIB d'ici à 2022. » Monsieur le ministre Darmanin, ma question est simple : qu'avez-vous à répondre aux critiques avisées de ces experts indépendants ?

Vous nous interrogez plus particulièrement sur la question des effectifs de la fonction publique. Elle accompagne la modernisation que nous menons dans chaque domaine. Nous travaillons là aussi avec une ligne de conduite : garantir la qualité des services qualité des services et rapprocher, à chaque fois que nous le pouvons, les services publics des usagers. Nous défendons ensemble un de géographie revisitée, pour faire en sorte qu'il y ait plus de points de contact, notamment en matière de finances publiques. Nous travaillons avec le ministère de la cohésion des territoires pour développer une offre de services de qualité dans les maisons de services au public. Notre objectif

de vos efforts en matière de réduction du déficit. J'ai consulté les 48 fiches relatives à la mise en oeuvre des réformes prioritaires du Gouvernement. J'y ai lu des choses intéressantes, mais je n'y ai vu nulle part une réduction de la dépense publique. Il faut aller plus vite

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Il y a quelques semaines, monsieur le ministre, je vous interrogeais sur l'interdiction des serres chauffées en agriculture biologique. Votre réponse m'avait alors paru ambiguë, et je vous l'avais fait savoir. Depuis, la Fédération des agriculteurs bio, les citoyens et les ONG se sont emparés de cette question avec force, notamment une pétition, qui a recueilli à ce jour plus de 80 000 signatures. Des distributeurs, et non des moindres, se sont engagés à ne pas vendre de produits bio récoltés sous serres chauffées. le journal publiait une tribune, signée par une centaine de parlementaires, vous appelant à prendre position en faveur de l'interdiction de la production bio à contre-saison. Cette mobilisation et sa forte médiatisation sont la preuve de l'attachement des acteurs de la filière bio et des consommateurs-citoyens au cahier des charges AB, garantie de qualité et de respect de l'environnement. de la réunion du Comité national de l'agriculture biologique, pouvez-vous nous dire si, comme le laissent penser vos dernières interventions dans les médias, vous soutiendrez une interdiction claire des serres chauffées en agriculture biologique ?

est de savoir dans quel cadre nous fixons les règles. C'est la ligne que j'ai fixée au Comité national de l'agriculture biologique, qui devra prendre une décision jeudi. Nous ne sommes pas opposés au chauffage des serres. Nous sommes contre la surtransposition

monsieur le ministre, c'est aux acteurs de prendre leurs responsabilités, mais la voix du Gouvernement, vous le savez bien, a une importance forte. Le cahier des charges de l'agriculture bio, élément de notre patrimoine national, est exigeant et cohérent. Il est important d'en préserver la qualité. Le bio- c'est son son essence -doit être local. Il doit respecter la saisonnalité et le lien au sol. Ouvrir la voie à l'industrialisation de ce label est un non-sens, à la fois sur le plan environnemental, à l'heure de l'urgence

Alors que notre pays est de plus en plus confronté aux tentatives de certains de remettre en cause les fondements mêmes de notre unité, en particulier la laïcité, nous avons appris par un journal de province, monsieur le aux préfets une circulaire pour accompagner l'émergence de structures départementales des acteurs du culte musulman, préfigurant ainsi la mise en place d'un maillage territorial, comme le souhaite l'association Musulmans de France, l'ancienne UOIF, dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle est la branche française des Frères musulmans. Si cette information est exacte, est-ce bien le rôle de l'État, des préfets, de s'immiscer dans l'organisation d'une religion, quelle qu'elle soit ? Si cette immixtion du représentant de l'État dans l'organisation d'un culte se confirme, vous engagez le pays dans un recul de la laïcité

Nombreux sont les citoyens de notre pays qui attendent une prise de parole claire du Président de la République et du Gouvernement sur ce sujet, sur les valeurs de la République et sur la laïcité. Il appartient à toutes les religions de se fondre dans la République, sans accommodement, et non l'inverse. La loi de la République est au-dessus de la foi pour chacun d'entre nous, quelle que soit sa religion. Les menaces qui pèsent sur la cohésion nationale sont réelles, monsieur le secrétaire d'État. Arrêtons de tolérer l'intolérable ! Cessons de céder aux pressions religieuses ! Pour faire appliquer tout cela, nul besoin de réunion chez le préfet, il faut simplement du courage politique et la volonté de refuser toutes les pratiques religieuses qui mettent à mal notre liberté et la neutralité de l'État. Entendez, monsieur le secrétaire d'État, le cri d'alarme de l'Association des femmes élues de l'Isère, entendez le cri de femmes courageuses qui s'appellent Zineb, Zohra, Fatiha ... Votre responsabilité est de ne jamais laisser vaciller la République et la laïcité

pour exprimer non seulement leur lassitude, mais aussi leur colère risque de durer, alors que l'été est là, avec ses menaces de feux de forêt, rendues encore plus inquiétantes par les fortes chaleurs et la canicule. De plus en plus sollicités et trop souvent pour des missions qui ne correspondent pas à leurs compétences, confrontés à des manques d'effectifs et de moyens, ainsi qu'à de très nombreuses agressions, les pompiers doivent faire face à la disparition des services publics de proximité. C'est ainsi que, dans les zones rurales touchées de plein fouet par la désertification médicale, la situation devient particulièrement préoccupante. Les pompiers sont fréquemment appelés à remplacer les ambulanciers. Dans les départements de la Gironde et de la Dordogne, cette catégorie d'intervention a augmenté de 13 %, ce taux De 2003 à 2018, le nombre d'interventions annuelles effectuées par les pompiers est passé de 3,5 millions à 4,6 à 4,6 millions. Le département de la Gironde a subi une hausse de 16 %, celui des Landes de 26 %. Cette année, la Gironde prévoit de dépasser le seuil des 140 000 interventions, contre 115 000 en 2017. de l'activité opérationnelle ne peut se compenser par une rationalisation et une mutualisation des moyens, dont les limites inquiètent à juste titre toute une profession.

d'assurer la protection des pompiers et la nécessaire coordination avec les autres acteurs de la sécurité sur l'ensemble des territoires. Monsieur le secrétaire d'État, quelle réponse avez-vous l'intention d'apporter aux pompiers, qui n'en peuvent plus ? Il y a véritablement urgence ! La parole est

dans le cadre de protocoles départementaux pour mieux lutter contre ce phénomène, d'abord en organisant l'action coordonnée des secours et des forces de l'ordre, puis en assurant une plus grande communication sur la prévention de nos sapeurs-pompiers. Une grande campagne est prévue à l'automne 2019 sur ce sujet.

Croyez bien, monsieur le sénateur, que nous sommes très déterminés à soutenir l'action des sapeurs-pompiers, dont je veux ici, devant le Sénat, de nouveau saluer l'engagement, le courage, la détermination et le grand professionnalisme. Avant de poursuivre notre

Nous devons donc trouver un panel de solutions pour lutter contre toutes ces causes, qui sont extrêmement diverses. Il existe en fait une distorsion à l'échelon mondial entre l'offre et la demande, car la demande est croissante dans tous les pays émergents.

qui sont très difficiles à obtenir, car très difficiles à produire. Nous nous efforçons également de renforcer la capacité de régulation des pénuries par l'Agence de sécurité

Concernant l'homéopathie, vous aurez ma réponse demain, monsieur le sénateur.

soixante jours pour officialiser, pour graver dans le marbre le paiement d'une subvention qui est due,

Dans l'immense majorité des municipalités, notamment dans les petites et les moyennes communes, tout se passe bien. Je ne suis en revanche pas sûr que, dans toutes les grosses collectivités, en particulier dans les EPCI, la fluidité soit de même nature que dans les communes moyennes.

c'est celui qui va recevoir l'argent qui envoie une facture alors que, dans le cas présent, c'est celui qui décide de donner de l'argent qui envoie le document qui déclenche le versement. Techniquement, le rapprochement avec la commande publique est, à mon avis, un petit peu scabreux.

L'article 788 du code général des impôts offre à tout ayant droit redevable des droits de mutation par décès la possibilité, en accordant un don à un organisme reconnu d'utilité publique, dans les six mois du décès, de réduire d'autant le montant de son imposition successorale. Dans les faits, ce délai de six mois est trop court pour la réalisation à titre définitif de la libéralité, même lorsqu'il s'agit d'un don en espèces. le donateur potentiel n'a pas nécessairement une connaissance immédiate de sa qualité d'héritier, de l'existence de l'avantage fiscal auquel il peut prétendre ou même, parfois, des disponibilités successorales. Je propose donc de prévoir l'allongement de ce délai de six à douze mois afin de faciliter les dons sur les successions. Je suis bien conscient que cette proposition aurait plus sa place dans une loi de finances, mais elle vise également à améliorer la trésorerie des associations. Son adoption permettrait d'augmenter

L'article L. 612-4 du code de commerce dispose que toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe.

pour garantir un véritable contrôle. Tracfin propose de le supprimer et de le remplacer par un audit légal spécifique intégrant les vigilances Lutte contre le blanchiment et Financement du terrorisme, qui pourrait être défini et appliqué dès le premier euro d'argent public versé ». J'entends déjà les commentaires et les cris d'orfraie pour évoquer les joueurs de boules

tenue de la comptabilité et la publicité qui en est faite, afin de mieux respecter les exigences en matière de transparence sans pour autant alourdir le formalisme demandé aux associations.

attention. Par ailleurs, une partie de cet amendement est satisfaite par les dispositions légales actuelles, puisque la tenue de comptes annuels est aujourd'hui une obligation, y compris pour ces associations. Quant aux autres questions, je prendrai connaissance avec attention des travaux qui seront menés au Sénat.

s'inspirant de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique et des textes encadrant les associations

des conséquences très importantes sur l'organisation historique des cultes en France et des associations qui concourent à l'exercice de cette liberté publique.

de grandes conséquences. C'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai sur cet amendement.

La parole est à Mme Maryse Carrère. Comme l'illustre la rédaction des articles 2 et 4 de cette proposition de loi, l'article 200 du code général des impôts présente une importance particulière dès lors que, au-delà des exonérations fiscales qu'il permet, son champ d'application sert également de référence pour l'application d'un certain nombre de dispositions relatives aux associations.

200, elle bénéficie aux associations non cultuelles comme cultuelles. C'est par exemple le cas de l'article 2, qui ouvre le droit à un prêt inter-associations, ou de l'article 4, qui permet à l'État de confier à des associations la gestion de biens immeubles dont il est devenu propriétaire à l'occasion d'une instance pénale. Cet amendement Cet amendement vise donc à évaluer la portée financière des ambiguïtés et les incohérences découlant de toutes les dispositions postérieures à la loi de 1905 qui entrent directement en contradiction avec son article 2, lequel prévoit que la République ne subventionne aucun culte- cette disposition a également valeur constitutionnelle. Comme le soulignent les auteurs de la proposition de loi dans l'exposé des motifs, la part des exonérations fiscales dans le budget des associations est devenue supérieure à celle des subventions. Cela s'applique aussi aux associations cultuelles. Ainsi, afin de préparer une clarification plus vaste des régimes entre les associations de type loi 1901 et celles de type loi 1905, cet amendement vise à introduire la liste et l'objet de toutes les associations demandant à bénéficier de l'exonération prévue à l'article 200 des impôts dans les annexes annuelles au projet de loi de finances, afin de mesurer la part des associations cultuelles au sein de celles-ci.

Or il apparaît que ce régime n'offre pas de garanties suffisantes concernant l'usage à venir de ce mode de paiement, même si ces dons sont limités à 300 euros par mois et par numéro.

De telles opérations auraient dû faire l'objet d'une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, plutôt que de bénéficier de ce régime allégé. Cette disposition a modifié la loi de 1905, qui établit la séparation des Églises et de l'État et qui reste un texte constitutif de notre République. Cette modification de la loi de 1905 aurait mérité

amendement vise à ouvrir de nouvelles voies de financement aux associations. Aujourd'hui, le code électoral permet à un candidat, lorsque celui-ci a recours à une association de financement électoral, de reverser l'excédent qui figure sur son compte de campagne à une association de financement politique ou à un établissement reconnu d'utilité publique. La notion d'établissement reconnu d'utilité est trop restrictive. Nous proposons donc d'élargir la liste des organismes bénéficiaires de cet excédent à tous ceux qui sont visés à l'article 200 du code général des impôts. Ainsi, un candidat, une fois les élections passées, pourra par exemple reverser l'excédent de son compte de campagne à des oeuvres ou à des organismes d'intérêt général présentant un caractère philanthropique, éducatif, social, humanitaire ou encore lié à la défense de l'environnement. Cette disposition vise à ajouter de la souplesse à notre droit et permet de diversifier les sources de financement des associations,

Cet amendement a pour objet d'élargir la liste des associations pouvant bénéficier d'excédents du compte de campagne lorsque le candidat a eu recours à un mandataire personne physique.

qui prévoit la possibilité pour les parlementaires de siéger au sein des collèges départementaux du Fonds de développement de la vie associative, sur le modèle des collèges existant aujourd'hui pour la DETR. La parole est à

et qui ne devraient se mêler que de ce qui se passe en séance ! Non, la crise des « gilets jaunes » et les revendications des citoyens, qui ont eu beaucoup d'échos ces derniers mois, montrent que l'on a besoin de cette proximité. L'élu doit être au plus près de tout ce qui

vous avez contesté par cette loi la légitimité des élus du peuple. Pensez-vous que cette légitimité soit moindre que celle d'un fonctionnaire de l'État que vous nommez ? Je ne la remets pas en cause, mais je considère que, en exigeant, par cet amendement, que tous les parlementaires intéressés siègent dans cette commission, nous faisons ici oeuvre utile pour notre démocratie.

Au travers de la question de notre collègue apparaît le souhait légitime de savoir, d'être informé et d'être associé. La réserve parlementaire, à qui on a attribué beaucoup de maux, était, il faut l'affirmer,

L'article 4 prévoit de façon très intelligente que puissent être mis à la disposition des associations les biens immobiliers saisis par l'État dans le cadre de procédures judiciaires. Cette volonté n'est absolument pas remise en cause pour toutes les associations cultuelles. Toutefois, par cohérence avec le régime particulièrement complexe et précis des biens immobiliers mis à disposition des cultes prévu par la loi de 1905, nous demandons que les associations cultuelles soient exclues du périmètre de l'article 4,

aux associations concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement, nous paraît inadaptée. Si les associations régies par la loi de 1901 peuvent relever de ce champ, d'autres relèvent également de cette catégorie, notamment des sociétés commerciales. L'ajout de cette disposition, par un amendement de Mme la rapporteur, aura des conséquences bien plus larges que l'objet de la proposition de loi, qui vise les seules associations. Aussi, je m'interroge sur la réelle portée et la place de cette mesure dans ce véhicule législatif.

L'ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations avait exclu les biens de ces dernières du champ du droit de la préemption urbaine. Or la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a réécrit l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme avec, pour effet involontaire, de faire disparaître cette mesure et de soumettre de nouveau ces biens au droit de préemption. Lors de la première lecture du projet de loi, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteur visant à réinstaurer cette exonération des biens des associations du régime de préemption. L'article 4 corrigeait simplement les effets de cette suppression malencontreuse. cet article a été supprimé en commission sénatoriale au prétexte qu'il contrevenait au droit de regard des communes et instituait une restriction du droit de préemption des collectivités, déjà très encadré. Le Sénat, par cette suppression, entendait réaffirmer la priorité des projets publics sur tout autre, autorisant, pour ce faire, à user de la préemption sur tout bien. Il convient de rappeler que cet amendement ne visait qu'à qu'à rétablir l'exonération instaurée par l'ordonnance du 23 juillet 2015, mais dont l'article avait ensuite été censuré par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme que l'objet de cette mesure était d'accroître le financement du secteur associatif, de permettre à une fondation reconnue d'utilité publique à l'occasion de sa création de se constituer une dotation initiale ce type de libéralité et mutation d'immeuble à titre gratuit. Les donations constituent une source importante d'apports pour les associations et les fondations. À titre d'exemple, entre 2013 et 2015, 35 % des fondations créées reconnues d'utilité publique ont reçu une dotation composée de biens immobiliers issue d'une donation, pour une valeur globale allant de 500 000 euros à 17 millions d'euros. Dans de nombreux cas, les immeubles apportés à la dotation sont ceux qui permettent la réalisation de l'objet social de la structure. Pour les associations reconnues d'utilité publique, les donations constituées de biens immeubles ont représenté entre 2013 et 2015 respectivement 37,5 %, 53 % et 27 % des donations consenties. Face à ce constat, associé à celui de la raréfaction des financements publics, il apparaît pertinent de rétablir cette exclusion du champ d'application du droit de préemption des donations immobilières effectuées au profit des organismes non lucratifs de façon à maintenir la diversité et les possibilités des apports privés. C'est la raison pour laquelle nous soutenons que l'article 4 doit être réintroduit dans la proposition de loi.

qui avait pour objet de rendre inapplicable le droit de préemption aux immeubles cédés à titre gratuit à des fondations, des congrégations ou des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités.

nous paraissent manifestement inappropriées. Il ne s'agit pas d'opposer, d'un côté, le droit des collectivités territoriales et, de l'autre, le secteur associatif. Comme cela a été souligné, cette disposition, qui figurait dans la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, a été déclarée contraire à la Constitution pour des raisons de forme. Elle avait pour objet de corriger les contradictions apportées par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. En son temps, le Sénat avait adopté cette mesure sans modification lors de l'examen de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté précitée.

lequel est extrêmement complet. Il est publié et mis en ligne sur le site internet de cette association spécialisée dans le financement, la trésorerie et la fiscalité des associations. La ville de Bordeaux, par exemple, s'appuie sur les travaux réalisés par cette association nationale, mais elle n'est pas la seule : c'est sur cette étude que s'appuie Bercy chaque année pour la de surcroît largement commentée et relayée par la presse. C'est pourquoi, considérant que nous disposons de tous les outils et de l'expertise nécessaire, je vous propose d'adopter cet amendement de suppression de l'article.

à M. Joël Guerriau. Cet amendement a pour objet la réalisation d'un rapport pour déterminer notamment l'impact des mesures fiscales prises depuis la dernière élection présidentielle sur le budget des associations. En effet, les réformes fiscales de ces deux dernières années- suppression de l'ISF, réforme de la CSG, mise en place du prélèvement à la source -ont abouti à la réduction des dons aux associations et ont donc eu un impact négatif sur leur trésorerie. La réalisation d'un tel rapport permettrait d'en mesurer les principales causes de la manière la plus claire possible.

d'apporter des précisions quant aux modalités de l'appel de dons entraînant une obligation de déclaration préalable. L'appel à la générosité du public implique une action de sollicitation ayant pour contrepartie le versement d'un don en numéraire. On considère qu'il y a sollicitation active lorsqu'une association par exemple, un bouton « don » pratique également des actions de promotion de ce mode de collecte : mailing renvoyant vers le site, e-mailing renvoyant vers le bouton « don », mise en place de bandeaux publicitaires, etc. A l'inverse, l'envoi d'informations sur les modalités de versement d'un don lorsque le donateur en fait la demande ou bien un d'information sur le site internet dont prend connaissance la personne qui a décidé spontanément de visiter le site ne constitue pas une démarche de sollicitation active de l'organisme. Il s'agit d'un amendement de précision, qui, je le crois,

lors de la constatation du dépassement de ce seuil. En effet, il sera difficile, voire impossible de faire une déclaration préalable quand il s'agit d'un premier appel public ou lorsque le seuil est atteint pour la première fois en cours d'année. Cet argumentaire est très technique, mais il est sûrement très juste.

Selon l'IGAS, elles étaient 57 % à s'y conformer en 2012, 46 % en 2015 et seulement 39 % en 2017. Or la publication transparente de ces comptes est un objectif prioritaire de gestion des dépenses publiques, dès lors que les fonds publics représentent 49 % du financement des associations. Il s'agit également d'une obligation à l'égard des donateurs privés, qui sont en droit de connaître l'utilisation qui est faite de leurs dons.

Celle-ci martèle que « la publicité des comptes incluant le compte d'emploi des ressources, qui doit retracer spécifiquement l'emploi des ressources issues de la générosité, est une condition essentielle de la transparence ». Selon les chiffres déjà évoqués, 39 % des associations et fondations publient régulièrement leurs comptes sur le site de la DILA et 43 % si l'on compte celles qui le font sur leur propre site internet. Néanmoins, comme le note l'IGAS, 30 % des associations qui se soumettent à la publication le font de manière insatisfaisante, ne publiant pas le compte d'emploi des ressources, ou en publiant une version incomplète, ce qui réduit en réalité à 27 % le taux d'associations et de fondations en règle.

qui exercent leur activité dans le domaine de l'insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle. Or lorsqu'une association qui propose ce service, mais qui peut avoir d'autres activités, se transforme en fondation, la préfecture retire son agrément, alors même que la fondation souhaite poursuivre cette activité, au seul motif que le terme de fondation n'est pas expressément indiqué dans l'article L. 213-7 du code de la route. Les nouvelles fondations n'ont alors pas d'autre solution que de cesser leur activité d'enseignement, pénalisant ainsi un public souvent fragile, ou de créer une association, ce qui est souvent contraignant d'un point de vue tant administratif que financier et fiscal. Des associations devenues fondations sont aujourd'hui confrontées à ce type de situation. Ainsi, la fondation Massé-Trévidy, dans le Finistère, qui forme gratuitement chaque année 300 personnes au sein de sa structure « Roulez jeunesses », ne pourra plus proposer cette activité, faute d'agrément. D'autres fondations, comme les Apprentis d'Auteuil, pourraient également être concernées. C'est pourquoi, afin de faciliter l'activité d'enseignement de la conduite, il est proposé de compléter l'article L. 213-7 du code de la route en y incluant les fondations au sens de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987.

réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros au titre des services fournis en France, au sens de l'article 299 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi portant création

qui a été rendu public voilà quelques semaines à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une mesure de bon sens. Comme le dit Bruno Dalles, le directeur de Tracfin, si l'on adhère à une association, c'est que l'on adhère à son idéologie et à la cause qu'elle défend. Ce n'est pas exactement la même chose d'adhérer à la Société protectrice des animaux qu'à Génération identitaire.

Madame Goulet,

qui ont été déposés par les membres de notre groupe visant à clarifier la différence des règles financières devant s'appliquer, d'une part, aux associations cultuelles et, d'autre part, aux associations non cultuelles. Trop souvent, en effet, nous observons une attitude ambiguë à l'égard du principe de laïcité : d'un côté, l'union nationale pour en glorifier le principe et, de l'autre, des contradictions au moment de sa mise en oeuvre. Concernant la relation financière entre l'État et les cultes, la loi de 1905 est parfaitement claire, et toutes les entreprises visant à atténuer les dispositions de son article 2 nous semblent de nature à l'affaiblir. C'est pourquoi nous souhaitons symboliquement inscrire dans l'intitulé